Monsieur le président,

soit 607 millions d'euros. Cette hausse est supérieure de 200 millions d'euros à la trajectoire prévue par l'article 1 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Toutefois, hors les mesures de périmètre et de transfert intervenues depuis le vote de cette loi, l'écart avec celle-ci n'est que de 100 millions d'euros. Cet effort budgétaire représente ni plus ni moins qu'une hausse nécessaire des moyens consacrés à l'exercice de cette mission régalienne. d'autant plus nécessaire que, l'an passé, le budget proposé n'était pas conforme à la trajectoire de la loi de programmation : l'augmentation était deux fois inférieure à l'annuité adoptée par le Parlement, pourtant quelques mois plus tôt Le budget qui nous est proposé constitue donc un rattrapage indispensable, car la situation demeure fragile, comme en témoigne la dégradation des principaux indicateurs de performance de la mission, notamment les délais moyens de traitement des procédures pénales ou civiles.

Les créations d'emploi sont marquées par la priorité stratégique fixée pour le budget pour 2021 du ministère : le renforcement de la justice de proximité, destiné à lutter plus efficacement contre la petite délinquance du quotidien. Ainsi, sur les 318 postes créés pour la justice judiciaire, 150 seront affectés au renforcement de l'équipe autour du magistrat. Tous les programmes de la mission sont concernés par cette priorité, mais la justice judiciaire figure en première ligne. En effet, les crédits alloués aux frais de justice augmentent de 127 millions d'euros, dont une partie renforcera les moyens d'enquête et d'expertise de la justice. Cette hausse répond à la technicisation croissante des enquêtes, mais constitue surtout une mesure de sincérité budgétaire, car ce poste à fait l'objet d'une sous-budgétisation récurrente ces dernières années. 15 millions d'euros supplémentaires sont alloués aux délégués du procureur, qui apportent une réponse pénale rapide dans les faits de délinquance du quotidien. Un effort particulier est consacré aux dépenses d'investissement : 164 millions d'euros de crédits supplémentaires sont accordés à l'administration pénitentiaire au titre du programme immobilier pénitentiaire, 270 millions d'euros sont consacrés au financement des 7 000 places qui seront créées d'ici à la fin du quinquennat et 25 millions d'euros aux études des opérations de la seconde phase de construction de 8 000 places supplémentaires, qui seront lancées d'ici à 2022. Par ailleurs, la transformation numérique du ministère se poursuit et prend tout son sens dans le contexte de la crise sanitaire. Dans cette perspective, 207 millions d'euros sont consacrés au plan de transformation numérique du ministère, qui s'accélère, s'agissant tant de l'équipement des juridictions en matériels que du développement de projets applicatifs. Ces investissements coûteux nécessitent toutefois un suivi attentif, afin que les délais soient respectés, mais surtout qu'ils soient utiles aux professionnels. Je terminerai par deux remarques à propos de la hausse de 28 millions d'euros des moyens consacrés à l'aide juridictionnelle, un effort qui intègre une enveloppe de 25 millions d'euros destinée à financer les mesures retenues par le Gouvernement à la suite de la mission confiée au printemps dernier à Dominique Perben au sujet de l'avenir de la profession d'avocat.

cette réforme, notamment la revalorisation de l'unité de valeur, est traduite dans l'article 55 , rattaché à la mission « Justice », adopté à l'Assemblée nationale par la voie d'un amendement du Gouvernement. Nous ne disposons d'aucune évaluation préalable de l'article, puisque cette réforme ne figurait pas dans le projet

avis. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, voilà plusieurs années que la commission des lois plaide en faveur d'un renforcement substantiel des moyens de la justice, notamment de son administration pénitentiaire,

Cette augmentation importante ne nous paraît pas excessive au regard de l'ampleur des besoins en matière de personnel, d'entretien des locaux et de construction de nouvelles places de prison. Ces moyens supplémentaires doivent permettre de financer les deux priorités de l'administration pénitentiaire

Enfin, plus de 400 créations de postes sont prévues pour constituer les équipes ayant vocation à travailler dans les futurs établissements pénitentiaires. a pour ambition de réduire la surpopulation carcérale en construisant de nouvelles maisons d'arrêt et de favoriser la réinsertion en créant des structures d'accompagnement vers la sortie, les SAS, et en expérimentant des établissements tournés vers le travail. Actuellement, 654 places sont en cours de réalisation, et un marché a été notifié aux entreprises pour 3 450 places supplémentaires. L'an prochain, deux établissements devraient être livrés, à Lutterbach, près de Mulhouse, et à Koné, en Nouvelle-Calédonie. L'ouverture de ce dernier établissement améliorera la qualité d'un parc pénitentiaire souvent fort dégradé dans nos départements et collectivités d'outre-mer. L'année 2020 a été marquée par une forte baisse de la population carcérale, consécutive à la crise sanitaire, qui pourrait nous conduire à nous interroger sur la pertinence de maintenir ce programme immobilier il est vraisemblable que le nombre de détenus va rapidement retrouver son niveau habituel, maintenant que les juridictions ont repris leur activité. De plus, la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de cassation, puis du Conseil constitutionnel, sur la notion de conditions indignes de détention constitue une incitation supplémentaire à investir dans nos prisons. Nous devons faire disparaître ces situations choquantes, où trois personnes partagent une cellule de neuf mètres carrés avec un matelas au sol, si nous voulons éviter que des juridictions décident de libérations inopportunes du point de vue de la politique pénale ou de la sécurité publique.

d'autant que cette augmentation est supérieure de 200 millions d'euros à l'annuité 2021 prévue par la loi de programmation du 23 mars 2019 et même conforme à la trajectoire votée par le Sénat.

En effet, à la lumière de la réalité de la vie des tribunaux et des justiciables, les moyens accordés sont à relativiser, compte tenu des retards accumulés dans les investissements en matériel, les recrutements et le paiement de charges antérieures.

En effet, sur ces 1 082 emplois, seuls 168 sont pérennes- 50 magistrats, le reste pour les greffes -, soit moins que les 513 emplois pérennes créés en 2020. Si le taux de vacance des magistrats est aujourd'hui de moins de 1 %, celui des greffiers avoisine les 7 %, avec 670 emplois vacants. La promesse de résorber la vacance d'ici à la fin de 2021 est donc loin d'être tenue. Par ailleurs, les 914 recrutements contractuels- juristes assistants et aides-greffiers, qualifiés de « sucres rapides » -sont destinés à résorber les difficultés des juridictions pénales de proximité. Favoriser la justice de proximité est louable, mais la vraie justice de proximité, celle du quotidien, celle qui concerne tous les citoyens, est la justice civile ; la justice pénale, elle, ne concerne que les délinquants- d'ailleurs, elle traite trois fois moins d'affaires que les juridictions civiles. civiles. La courbe des stocks des tribunaux judiciaires est alarmante. L'intégration des juridictions de la sécurité sociale a importé plus de 200 000 affaires en attente, et la crise sanitaire et la grève des avocats ont alourdi ce stock de plus de 18 000 affaires, alors même que le nombre de nouvelles affaires a baissé de 39 %.

nous, le budget ne va pas assez loin dans cette direction. Prévues à hauteur de 27,5 millions d'euros en 2021, les augmentations coûteront 50 millions d'euros en année pleine, soit bien moins que les 100 millions d'euros recommandés par la mission Perben afin de relever l'unité de valeur à 40 euros, comme les professions le demandent.

appartenez ; utile encore lorsqu'il permet au tribunal de Bobigny d'être hors d'eau et à d'autres d'être câblés ou bien aménagés pour accueillir les justiciables.

Heureusement que, dans cet hémicycle, nous avons majoritairement dépassé les cinquante ans ... Sinon, nous ne comprendrions même pas ce que je vais vous dire. Figurez-vous, mes chers collègues, que certains applicatifs de la justice tournent encore sous Windows 3 et avec WordPerfect

un grand plan de rénovation numérique a été mis en place, d'un montant de 530 millions d'euros, dont 350 millions d'euros, soit près de 67

Bref, la justice n'est pas, techniquement, entrée dans le XXI siècle ! Monsieur le garde des sceaux, si l'on veut penser la justice et lui donner la force qu'elle mérite,

avis. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il m'appartient de vous présenter les crédits du programme « Protection judiciaire de la jeunesse », sur lesquels la commission des lois a émis un avis favorable. La protection judiciaire de la jeunesse représente 9,4 % des crédits de l'ensemble de la mission « Justice », moins d'un quart des crédits du programme « Administration pénitentiaire » et un peu plus d'un quart de ceux du programme « Justice judiciaire Les missions dévolues à la PJJ, qui assure le suivi de près de 150 000 jeunes chaque année, justifient qu'un examen spécifique de ses crédits et de ses missions soit réalisé chaque année par la commission des lois. Le projet de loi de finances pour 2021 dote la protection judiciaire de la jeunesse d'un budget de 789,8 millions d'euros hors pensions, en augmentation de 53,2 millions d'euros, soit 7,2 %, par rapport à la loi de finances initiale pour 2020. Cette augmentation particulièrement importante est supérieure à celles des années antérieures ; elle est en rapport avec la hausse de l'ensemble de la mission, mais doit être soulignée et saluée. Toutefois, cette augmentation doit être analysée au regard de l'effet de rattrapage nécessaire à la concrétisation des engagements des années antérieures en matière de créations de postes et des enjeux d'adaptation importants auxquels fait face la PJJ, principalement- mais pas uniquement -en lien avec la réforme de l'ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs, dont l'entrée en vigueur est désormais reportée au 31 mars Si le projet de budget pour 2021 prévoit de nouvelles créations de postes, la PJJ a souffert, au cours des dernières années, d'un écart croissant entre le nombre de postes théoriquement ouverts par le budget et une dotation en crédits insuffisante pour recruter effectivement des personnels au sein des différents cadres.

auquel la PJJ doit avoir recours ; ceux-ci constituent près de 19,7 % de ses effectifs. En l'état, le budget de la PJJ prévoit la création nette de 40 postes, dont 19 postes liés à l'ouverture de nouveaux centres éducatifs fermés et 20 postes pour la participation aux cellules de recueil d'informations préoccupantes. Un emploi sera créé pour le suivi des mineurs en milieu ouvert, vers lequel 83 emplois seront redéployés par ailleurs. Le renforcement et la formation des équipes d'éducateurs sont essentiels pour mettre en oeuvre le nouveau code de la justice pénale des mineurs. En l'état des stocks d'affaires et de l'organisation des services, la mise en oeuvre de la réforme au 31 mars prochain sera donc difficile. Un autre axe essentiel du budget la PJJ depuis deux ans est la création des centres éducatifs fermés. Déjà importante au regard du nombre de jeunes placés en leur sein, la part de ces structures dans les dépenses de la PJJ est amenée à croître, avec la création de vingt nouveaux CEF dans les prochaines années.

Nous allons connaître, à la suite de la crise sanitaire et sociale que notre pays vit, une multiplication des gens en grande pauvreté. La question

de professeurs de droit et d'éducateurs ont trouvé que la version de l'ordonnance ressemblait trop à la justice des majeurs. Il y a 850 mineurs incarcérés en France.

des mineurs délinquants était bénéfique pour la suite. Nous resterons pour notre part totalement fidèles à l'esprit de l'ordonnance de 1945 : le jeune doit d'abord être éduqué. Il faut s'en donner les moyens,

et que l'on s'occupe davantage de leur travail, de leur santé, notamment psychiatrique, et de leur insertion à la sortie pour éviter les sorties sèches, qui sont tout à fait négatives.

de déposer un texte de loi d'ici au mois de mars. Nous savons que vous y travaillez en préparant un amendement

au sein de notre appareil judiciaire. Durant le premier confinement, l'essentiel du contentieux civil a en effet été abandonné. Le contentieux pénal, lui, a été maintenu, mais dans des conditions dégradées en raison du recours à des dispositifs défavorables aux prévenus. Il va sans dire que les garanties accordées aux justiciables s'en sont trouvées détériorées. Face à cette situation, notre nouveau garde des sceaux avait promis un « effet Dupond-Moretti » sur le budget de la justice. Nous constatons effectivement une augmentation de 32 % des moyens accordés à cette mission, à hauteur de 12 milliards d'euros en autorisations d'engagement. Nous accueillons favorablement cette nouvelle. Dans les faits, cependant, il convient de rappeler que cette hausse importante est principalement due à un rattrapage lié au retard pris par le PLF pour par rapport aux objectifs fixés par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice votée en 2019. Par ailleurs, malgré ces chiffres encourageants, la France reste l'un des mauvais élèves de l'Union européenne en matière de budget accordé à son système judiciaire. Notre pays compte trois procureurs pour 100 000 habitants, contre douze dans les États membres de l'Union européenne. De même, avec un budget de 5,6 euros par habitant consacré à l'aide juridictionnelle, la France se situe au-dessous de la moyenne européenne, qui est de 6,5 euros. Les exemples sont multiples et démontrent les carences de notre système de justice. Il est évident que les crédits accordés à cette mission ne sauraient combler le retard pris sur nos partenaires européens pendant des décennies. Pour autant, nous notons les éléments positifs de la mission « Justice » de ce PLF. Outre l'augmentation des moyens alloués à cette mission, les 2 450 emplois ouverts pour le fonctionnement de notre système judiciaire sont les bienvenus. De même, la hausse des crédits du programme « Justice judiciaire » devrait permettre de désengorger les tribunaux, tendant ainsi à garantir une justice de proximité effective pour nos concitoyens. nous nous montrons plus réservés quant aux sommes attribuées à l'ouverture de 15 000 nouvelles places en milieu carcéral. Nous sommes évidemment favorables à l'encellulement individuel des prisonniers. Nous saluons donc les décisions prises par votre prédécesseure Nicole Belloubet visant à remettre en liberté des détenus en fin de peine. Cependant, constaté que la tendance est davantage au « tout carcéral ». Ainsi encourageons-nous le Gouvernement à favoriser le recours accru aux peines alternatives pour les petites peines. Nous sommes convaincus que le garde des sceaux, avocat pénaliste, sera sensible à cette thématique. Je souhaite conclure cette intervention en mentionnant les crédits alloués au programme « Protection judiciaire de la jeunesse ». Ce budget prévoit notamment l'ouverture de cinq nouveaux centres éducatifs fermés. Nous tenons à rappeler que nous sommes défavorables à l'enfermement de mineurs sans encadrement adapté.

de l'enfance. La justice des jeunes devrait favoriser leur éducation et leur réhabilitation plutôt que leur répression. les progrès notables réalisés dans ce budget. Ouh là ! Cet effort doit être soutenu, et il est nécessaire que la dynamique enclenchée s'amplifie dans les années à venir.

Ces crédits permettront de rattraper et même de dépasser les prévisions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en deçà desquelles nous étions l'année dernière. Ils aideront aussi et surtout à mettre en oeuvre les priorités du Gouvernement pour la justice de notre pays, priorités, monsieur le garde des sceaux, que vous avez souhaité accorder à la justice de proximité et à l'accès au droit ainsi qu'à l'administration pénitentiaire. Dans le bleu budgétaire, la justice de proximité est définie comme « celle du quotidien des justiciables, dont l'ambition est, d'une part, de lutter plus efficacement contre la petite délinquance du quotidien, au plus près des victimes et, d'autre part, de renforcer l'action judiciaire de proximité par un rapprochement, au plus près des territoires, Cela passe donc par un renforcement important des moyens humains. Ce budget permettra de procéder à 1 500 recrutements nets au cours de l'année qui arrive, 240 de plus que ce que la loi de programmation prévoyait. À ces recrutements s'ajouteront 950 emplois supplémentaires inscrits en fin de gestion pour l'année 2020. Cela passe aussi par la mise en oeuvre du plan de transformation numérique. La crise sanitaire que nous traversons nous a montré combien celui-ci était un enjeu majeur pour la justice de notre pays. Je sais que des investissements considérables ont d'ores et déjà été engagés. Cependant, lors d'un déplacement au tribunal de Paris le 19 novembre dernier, une délégation de la commission des lois à laquelle j'ai participé a pu constater qu'il fallait continuer de mettre l'accent sur l'équipement numérique et investir dans des logiciels plus modernes. L'accès aux droits des citoyens les plus en difficulté contribue également à cette justice de proximité. Aussi, je voudrais saluer l'effort budgétaire de 55 millions d'euros consacré à l'aide juridictionnelle, prévoyant une revalorisation de la rétribution des avocats, qui font un travail remarquable au profit de cette catégorie de citoyens. Il s'agit- vous l'avez rappelé, monsieur le garde des sceaux -d'une première avancée pour atteindre l'objectif de 96 millions d'euros fixé par la mission Perben et recommandé par nos collègues députés Naïma Moutchou et Philippe Gosselin.

je vous ai interrogé sur le problème que constitue, en matière de proximité de la justice, l'éloignement du justiciable mahorais de son juge d'appel, situé à La Réunion. Je concède qu'il s'agissait peut-être d'une manière un peu rude de vous accueillir, alors que vous veniez d'être nommé au Gouvernement, et j'en suis désolé. Mais, têtu comme je suis, je reviens à la charge et souhaiterais qu'on puisse trouver ensemble une solution acceptable à cette situation unique dans toute la République. L'histoire, la culture, l'état de développement des deux départements de l'océan Indien ne sont pas les mêmes. Le procureur général, pour ne prendre que cet exemple, officie à 2 000 kilomètres de Mamoudzou, dont la chambre détachée fonctionne comme un satellite de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Comment peut-il décider efficacement de la politique pénale de ce territoire s'il n'en connaît pas empiriquement la réalité ? Enfin, ce budget consacre un effort important en matière d'investissements immobiliers, en particulier en faveur de l'administration pénitentiaire. Certains voient dans la construction de nouvelles places de prison une contradiction avec la volonté du Gouvernement de réduire la population carcérale. En réalité,

Vous le savez, cette surpopulation est particulièrement préoccupante dans certains établissements ultramarins. C'est le cas au sein de mon territoire. Dans le contexte sanitaire actuel lié à l'épidémie de covid-19, la surpopulation carcérale est propice à la diffusion du virus. En juin dernier, 55 % de la population carcérale de la maison d'arrêt de Majicavo était testée positive. Ce budget ne permettra pas de régler toutes les défaillances de notre appareil judiciaire- c'est un fait mais il démontre la volonté du Gouvernement d'opérer un véritable changement. Il est important de souligner qu'il répond enfin aux attentes des citoyens et des acteurs de la justice, auxquels il apportera une véritable bouffée d'oxygène. Notre groupe est convaincu que ces crédits s'inscriront dans la durée. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez compris, il ne se privera pas de les voter avec enthousiasme. La parole est

En soi, nous ne pourrions que nous en réjouir, mais qu'en est-il vraiment d'un point de vue purement comptable et du point de vue de la répartition de ces crédits, autrement dit de ce qu'ils financent

que l'augmentation continue des moyens depuis 2012 est insuffisante pour sortir la justice de la pénurie à laquelle elle est confrontée. La comparaison avec nos voisins européens est à ce titre assez assez douloureuse : la France consacre moins de 70 euros par an et par habitant à son système judiciaire, quand l'Allemagne y consacre 122 euros, l'Autriche 107 euros et l'Espagne 79 euros. En parallèle, la France compte toujours deux fois moins de juges que la moyenne européenne pour 100 000 habitants. En outre, la période de confinement a mis en relief l'indigence du ministère de la justice, en particulier son sous-équipement structurel en matière numérique. Pis encore, la majorité du contentieux civil a été abandonnée pendant cette période et le contentieux pénal qui a été maintenu dégradation des garanties accordées aux justiciables : juge unique, audience en visioconférence, voire par téléphone, procédure sans audience et jugement en l'absence des prévenus ou retenus faute d'extraction, publicité restreinte, voire parfois supprimée. En outre, que signifient les chiffres si ce n'est ce qu'ils servent ? En l'occurrence, le premier poste budgétaire de la mission « Justice » demeure l'administration pénitentiaire, dont les crédits représentent plus de la moitié de l'enveloppe. l'Observatoire international des prisons souligne régulièrement l'inefficacité de l'augmentation du parc carcéral pour répondre à la surpopulation carcérale à laquelle nous sommes confrontés. Le deuxième poste budgétaire de la mission, la justice judiciaire, n'est pas sans poser problème non plus, puisque la mise en oeuvre de la réforme de l'organisation judiciaire se poursuivra en 2021. Rappelons que, par cette réforme, la carte judiciaire et les principes qui la gouvernent sont complètement bouleversés, ce qui marque un véritable tournant dans l'histoire de nos institutions judiciaires. La dualité tribunal de grande instance-tribunal d'instance disparaît au profit d'un tribunal judiciaire qui, par le biais d'une spécialisation accrue, instaure une hiérarchisation entre les juridictions d'un même département. Nous défendons au contraire une véritable justice de proximité, qui implique le maintien des tribunaux d'instance comme juridictions autonomes. Bien ancrés sur le territoire français, les tribunaux d'instance étaient vecteurs d'une justice de proximité. Ils traitaient la plupart du temps des contentieux concernant les plus faibles : mesures de protection, surendettement, crédit à la consommation, baux, litiges du quotidien ... Comment cette proximité avec les justiciables les plus précaires sera-t-elle maintenue ?

que le fond- l'accélération de la répression pénale, au détriment du temps éducatif de l'enfant -sont contestables. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas les crédits de cette mission, qui sont bien en deçà des moyens que nécessite le bon fonctionnement de ce grand service public qu'est la justice.

justice » au quotidien, non pas que nous nous désintéressions de tous les grands principes ni des sujets d'actualité, mais, dans le droit fil de l'avis budgétaire de ma collègue Dominique Vérien, je souhaite évoquer ces deux sujets

L'enjeu de la modernisation de la justice ne se limite pas à la seule question des infrastructures et du matériel, ni au nombre de milliers de portables qui seraient mis à sa disposition. Ce serait même à notre sens

Les trames d'actes sont rares et, me dit-on, peu mises à jour. Quant au logiciel civil, il n'est disponible à distance que pour un nombre limité d'utilisateurs. Au-delà de ce problème d'applicatifs,

au deuxième point de mon propos : la profession d'avocat, ô combien importante pour le bon fonctionnement de la justice. Comment donner aux avocats les outils leur permettant de réformer leur profession

Nous avons été stupéfaits, dans le cadre de la mission confiée par votre prédécesseur à Dominique Perben, de ne pas disposer de chiffres actualisés

doit nous conduire à poser de nouveau la question de l'expérimentation de l'avocat en entreprise. La profession n'a toujours pas trouvé sa position de cohérence en

avec votre ministère une convention globale. Cela permettrait certes de demander des augmentations de budget en matière d'aide juridictionnelle, mais aussi d'établir comment cette profession, en tant qu'auxiliaire de justice, peut contribuer dans les meilleures conditions à l'optimisation du système. La parole est

Boyer. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous pourrions nous féliciter de l'augmentation du budget en matière de justice et nous contenter de commenter les chiffres, mais nous devons aller plus loin qu'une considération arithmétique. Étudier le budget d'une mission, ce n'est pas seulement aligner des chiffres ; c'est aussi les analyser et les mettre en perspective. À la lecture du budget de la justice pour 2021, nous constatons, certes, une augmentation des crédits de près de 8 %. Nous notons aussi que leur montant, de 8,2 milliards d'euros, est effectivement supérieur de 200 millions d'euros au budget voté dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022

Si la loi de programmation prévoyait 8 milliards d'euros pour 2021, un retard de 115 millions d'euros a été enregistré en 2020. Je ne parlerai donc pas d'augmentation, mais de rattrapage budgétaire. Je pourrais aussi évoquer longuement les 15 000 places de prison qui devaient voir le jour pendant le quinquennat. Nous recensons 2 000 places construites. Pour obtenir les 7 000 places promises par le Gouvernement, il faudra attendre 2023. Ainsi, l'objectif des 15 000 places supplémentaires promises en 2017 ne sera pas atteint, loin de là. là. Au-delà du catalogue des promesses non tenues, c'est la dignité de l'accueil dans les prisons et la sécurité globale des Français qui me préoccupent aujourd'hui. En effet, comment lutter contre la récidive et le radicalisme si l'on ne construit pas de places de prison et si les agents pénitentiaires ne travaillent pas dans des conditions correctes ?

Par ailleurs, les quelques évolutions que l'on constate cette année apparaissent minimes au regard de ce qu'il reste encore à accomplir afin que la justice soit plus efficace, plus compréhensible et plus lisible pour nos concitoyens. Je crois, mes chers collègues, qu'il est impératif de continuer à renforcer davantage ce budget. La réforme de la justice des mineurs générera dans sa phase transitoire un surcroît de travail, de sorte que les besoins en personnels ne seront pas négligeables. L'extension, à moyens constants, de l'expérimentation de la nouvelle juridiction que sont les cours criminelles accaparera elle aussi des magistrats, des greffiers et des salles, au détriment au détriment d'autres activités, dont celles des cours d'assises qu'elles sont pourtant censées désengorger. Je rappelle d'ailleurs que près de 80 % des affaires de viol seraient requalifiées en « agressions sexuelles »- c'était l'esprit d'un texte ancien -pour rendre la justice plus rapide et désengorger les tribunaux. Dans son avis sur le viol et les agressions sexuelles publié en 2016, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes constate : « Le viol est un crime qui constitue la plus grave des violences sexuelles. Or il fait trop souvent l'objet de disqualification en agression sexuelle constitutive d'un délit. [ Si la disqualification n'a pas pour but de nuire aux intérêts des victimes, qui peuvent d'ailleurs s'opposer au renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, elle minimise la gravité du viol et remet en cause le principe d'égalité devant la justice. Le désengorgement des tribunaux, notamment des cours d'assises, ne doit pas se faire au détriment des victimes. Le viol est un crime, il doit être jugé comme tel. Enfin, la lutte contre les violences intrafamiliales, que vous avez déclarée priorité nationale, ne peut pas se contenter d'effets d'annonce. Vous savez tous que 146 femmes ont été tuées au sein de leur couple en 2019, soit vingt-cinq de plus qu'en 2018 ; vingt-sept hommes ont également été tués au sein de leur couple ; vingt-cinq enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents, dans un contexte de violences au sein du couple. Environ 143 000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré subir des formes de violence physique ou sexuelle, et des milliers d'autres ont été témoins de scènes de violence et en resteront sans doute marqués à vie. Derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle d'une souffrance insupportable et inacceptable. C'est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de l'implication de tous. Je présenterai différents amendements sur ce sujet. ce sujet. Nous devons renforcer la formation des policiers, des gendarmes et des magistrats. Interrogeons-nous encore sur l'accueil des victimes à tout moment de leur prise en charge. Renforçons les outils judiciaires de protection, tels que l'éviction du domicile des partenaires violents, l'ordonnance de protection et le téléphone grave danger. Les comparutions immédiates existent, mais restent insuffisamment utilisées. Améliorons le recueil des données par la justice en matière de violences conjugales : il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Améliorons les soins des victimes et développons les centres régionaux de psychotraumatisme. Prévoyons aussi davantage d'hébergements d'urgence et, surtout, sécurisons-les ! Enfin, donnons plus de moyens aux associations, que je veux remercier et saluer. Ces hommes et ces femmes font un travail remarquable pour les victimes. Mes chers collègues, nous pourrons éternellement faire voter des textes sur ces travées, mais ils resteront inapplicables si les finances ne suivent pas. Le combat contre les violences conjugales et pour la protection des enfants nous commande d'agir partout où la dignité, la morale et la loi l'exigent ! Nous devons le faire sans attendre Nous devons le faire sans attendre un nouveau budget. Le temps presse, et nous connaissons une grande partie des mesures qu'il faut prendre pour lutter contre ce fléau. Nous n'avons plus le temps d'attendre. II y a urgence pour les familles et pour les enfants que ces violences détruisent. Nous ne pouvons pas laisser plus longtemps les associations, les forces de l'ordre, les avocats et les magistrats pallier seuls les carences de notre législation. Le travail et le dévouement de ces hommes et de ces femmes forcent l'admiration et le respect. Pourtant, ils se sentent souvent livrés à eux-mêmes par manque de moyens, de temps ou de formation. Notre rôle de législateur est de les soutenir, possible, avant qu'ils ne se retrouvent dépassés par l'urgence. Au-delà des considérations budgétaires, je me permets de m'adresser à vous avec force, détermination et conviction, car être engagé dans la vie politique c'est avant tout défendre des convictions dans le cadre de l'intérêt général.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous avons le plaisir de saluer une hausse de 8 % du budget consacré à la justice pour l'année à venir. Cette mission en avait terriblement besoin, car les crédits qui lui sont consacrés n'avaient pas connu pareille augmentation depuis au moins La hausse prévue pour 2021 atteint les objectifs fixés par la loi de programmation ; elle les dépasse même de 100 millions d'euros. Cette trajectoire est la bienvenue au regard tant du rôle central de la justice dans notre pays que du manque chronique de moyens dont elle souffre depuis de trop nombreuses années.

L'augmentation du budget de la mission, cette année, est un signal encourageant. Nous espérons qu'il contribuera à recréer la confiance perdue. Aujourd'hui encore, la justice est trop lente, et pour cause En 2018, d'après la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, le nombre de juges professionnels par habitant, en France, était inférieur de moitié à celui de l'Allemagne. Il était même inférieur à celui de la Russie, de l'Ukraine ou encore du Kazakhstan.

Il est depuis peu repassé au-dessus. Il faut absolument en finir avec ce phénomène, car il est inacceptable qu'au pays des droits de l'homme des centaines de détenus dorment sur des matelas posés par terre. Nous avons besoin de plus de places dans nos prisons

Parallèlement, le développement des alternatives à la privation de liberté nous paraît judicieux. En les exacerbant, la pandémie a mis l'accent sur bien d'autres difficultés auxquelles l'institution judiciaire est confrontée en temps normal. Lors du premier confinement, nous avions appelé l'attention du Gouvernement sur le fait que certaines juridictions peinaient à continuer de travailler à distance, en raison notamment du manque de flexibilité des outils numériques. À ce titre, nous nous félicitons que le plan de transformation numérique soit poursuivi. Lorsque les circonstances l'imposent, il est indispensable que le travail de la justice puisse être effectué à distance, en toute sécurité. Nous remarquons cependant que de nombreuses solutions logicielles restent à finaliser. Par ailleurs, si certaines professions disposent du matériel nécessaire au travail à distance, d'autres, comme les greffiers, demeurent très majoritairement sans équipement. En plus d'être rapide, la justice doit être accessible. À cet égard, nous soutenons l'augmentation des crédits consacrés à l'aide juridictionnelle. Nous regrettons cependant qu'elle soit inférieure à celle qui est préconisée dans le rapport Perben. La hausse des crédits alloués à la justice, portée par ce projet de loi de finances, est un effort nécessaire. Les Français ont besoin de justice. Nous souhaitons que le budget pour 2021 soit l'amorce d'une nouvelle dynamique. Au-delà de ces quelques remarques, le groupe Les Indépendants soutiendra le vote

mes collègues l'ont déjà souligné, l'effort budgétaire global est important, à l'image des crédits du programme « Justice judiciaire ». Nous nous réjouissons tout autant des efforts en matière d'aide juridictionnelle que d'aide aux victimes. Il faut également apprécier la poursuite des créations de postes dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les juridictions pour mineurs. la réalité est aussi que ces hausses sont d'abord des efforts de rattrapage, après des années de sous-budgétisation catastrophique pour un service public aussi sollicité et fondamental pour notre pacte social. Il y a urgence, par exemple, sur la question des mineurs non accompagnés. Selon notre collègue Nathalie Delattre, on recense environ 3 000 MNA en Gironde, qui pâtissent de faibles mesures d'accompagnement et sont victimes de réseaux bien structurés. Or une explosion du nombre d'agressions et de manifestations de violences a depuis été observée localement, tandis que la question de la réponse pénale apportée pour assurer une certaine tranquillité publique se pose encore.

Dans le temps qui m'est imparti, je voudrais appeler votre attention sur une question spécifique, qui, loin d'être anecdotique, cristallise une forme d'insuffisance persistante des crédits alloués à la justice pour nos établissements pénitentiaires. Je parle des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, ces services déconcentrés de l'administration pénitentiaire départementale qui assurent le contrôle et le suivi des personnes condamnées dans leur parcours d'exécution des peines.

Or le travail des SPIP est rendu plus difficile, non seulement en raison des contraintes liées à la pandémie, le virus imposant de limiter les contacts physiques, mais aussi à cause du désengorgement des prisons, décidé par votre prédécesseur, afin d'éviter une trop forte contamination en milieu carcéral. Le nombre des personnes à suivre a considérablement augmenté, de sorte que les services peinent à tenir le rythme imposé. De telles circonstances auraient dû conduire à une augmentation significative des moyens et des effectifs. Or, sur ce point, le compte n'y est pas : les dépenses sont stables pour l'année 2021 à 42,5 millions d'euros,

le développement des autres types d'accueil et du secteur ouvert. Vous l'aurez compris, monsieur le garde des sceaux, les promesses de chiffres, certes encourageants, appellent désormais une mise en oeuvre rapide et efficace pour la société. Sous ces réserves, le groupe du RDSE votera ces crédits.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la justice consiste à organiser la vie en société : cette institution doit protéger les plus faibles et sanctionner ceux qui ne respectent pas le contrat social.

Souvent décriée, la prison reste la solution préconisée dans de nombreux cas. Même si les magistrats souhaitent trouver d'autres alternatives, elle reste pour l'instant incontournable, faute de mieux. J'aimerais m'attarder sur les multiples difficultés rencontrées par notre institution pénitentiaire et les agents qui la composent, aggravées encore depuis la crise sanitaire. La surpopulation carcérale atteint des sommets. Si le principe de l'encellulement individuel avait été proclamé dès 1875, puis réaffirmé en 2009, il n'a dans les faits jamais été appliqué. Le taux d'occupation des établissements pénitentiaires s'élevait à 116 %, au 1 janvier 2020, d'après la section française de l'Observatoire international des prisons. Cela signifie que la France compte plus de 70 000 prisonniers pour 61 000 places. Or cette surpopulation se concentre principalement dans les maisons d'arrêt destinées à accueillir les individus condamnés à de courtes peines de prison ou se trouvant encore en attente de leur jugement. Dans ces établissements, qui représentent environ les deux tiers de la population carcérale, le taux d'occupation moyen grimpe jusqu'à 138 %. Deux à trois individus sont donc contraints de partager la même cellule et dorment, très souvent, sur des matelas installés par terre. De telles conditions de détention rendent la surveillance des détenus plus ardue, voire inapplicable dans certains cas. Elles favorisent l'émergence de mutineries, permettent la prolifération de certaines maladies contagieuses et facilitent la constitution de réseaux criminels au sein même des établissements pénitentiaires.

face à leur incapacité à mener les missions qu'ils jugeaient nécessaires pour rétablir l'ordre dans les prisons et en assurer une gestion saine, tant pour eux que pour les individus incarcérés.

Ne nous voilons pas la face : une telle mesure ne sera efficace, sous réserve que les places promises soient bel et bien construites, que dans quinze ans, soit le temps que les infrastructures sortent de terre. Or le besoin de lutter contre la surpopulation dans les prisons est immédiat. Plus nous retarderons l'échéance, plus la situation sera dégradée, alors qu'elle est déjà au bord de l'implosion. Le Gouvernement, qui semble avoir pris la mesure de l'urgence, a décidé de privilégier les peines alternatives à l'enfermement. Dont acte ! Il faut désormais que l'exécutif se donne les moyens de ses ambitions. Adjointe à la sécurité de Tourcoing, avant mon élection au Sénat, j'avais mis en place des chantiers de travaux d'intérêt général, en relation avec les juges de l'application des peines du tribunal judiciaire de Lille. J'étais particulièrement satisfaite de proposer la remise en peinture de préaux d'écoles ou de salles de sport à des jeunes qui n'avaient jamais eu l'occasion jusqu'alors de montrer leur savoir-faire, même limité. Ces chantiers coûtent cher aux municipalités, car il faut prévoir du personnel d'encadrement. Il faut aussi convaincre les partenaires, très frileux à l'idée de recevoir des délinquants dans leurs structures. Monsieur le garde des sceaux, que prévoyez-vous pour développer ces prises en charge très difficiles à dénombrer ? Parmi les peines alternatives à l'enfermement, l'usage des bracelets électroniques peut-être envisagé pour surveiller les personnes condamnées hors des murs d'enceinte. Au-delà des stocks, a-t-on la certitude que les détenus libérés et placés sous le régime des bracelets électroniques seront bel et bien suivis par les services qui en ont la charge ? Ces services en ont-ils les moyens humains et matériels ? Encore une fois, rien n'est moins sûr ... Nos concitoyens sont inquiets en voyant le profil de certains détenus qui sortent de prison. Les services de renseignement ne seront-ils pas débordés compte tenu du nombre de ceux qui nécessiteront une surveillance accrue lorsqu'ils auront été relâchés dans la nature,

Qu'en est-il d'ailleurs des détenus dont on sait pertinemment que leur place se trouve davantage en hôpital psychiatrique qu'en prison ? Notre administration pénitentiaire est en fin de chaîne pénale, mais elle est essentielle pour assurer une réelle sanction et pour organiser la réinsertion des condamnés.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter le budget de mon ministère pour l'année 2021. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité des travaux et les échanges constructifs que nous avons eus lors de mon audition devant la commission des lois, le 17 novembre dernier. vous l'avez noté, ce budget permet à la fois le rattrapage de la loi de programmation pour la justice et le financement des priorités que j'ai affirmées au moment de ma prise de fonction, au premier rang desquelles la justice de proximité. C'est la première fois, en plus d'un quart de siècle, que le budget de la justice augmente autant, à hauteur de 8 % hors compte d'affectation spéciale.

607 millions d'euros supplémentaires, c'est-à-dire plus du double de l'augmentation votée en 2019 pour l'année en cours,

Ils viennent renforcer sans attendre les tribunaux, les établissements pénitentiaires et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse. Comme j'ai eu l'occasion de le dire devant la commission des lois, il ne s'agit pas de privilégier le contrat par rapport mais d'opter pour une réponse rapide- les « sucres rapides » -compte tenu de l'urgence qu'il y a à apporter un soutien immédiat au service public de la justice. Ces recrutements par contrat sont plus souples et plus rapides à mettre en place. Ainsi, pour renforcer les greffes, ils ne prévoient pas l'obligation du temps de formation de dix-huit mois à l'École nationale des greffes.

Madame le rapporteur pour avis Canayer, madame la sénatrice Benbassa, je vous le confirme, tous les métiers de la justice bénéficieront de ce plan de recrutement. Dans le détail, ce sont 1 100 emplois nets pour les tribunaux : 50 magistrats, 130 directeurs de greffe, 596 greffiers et renforts de greffe, qui viendront soulager sans attendre les juridictions en pourvoyant une partie des 700 vacances de postes de greffiers. 1 200 renforts pour l'administration pénitentiaire, dont 719 créations d'emplois de surveillants qui permettront de poursuivre la réduction du niveau de vacance des postes de surveillants, 335 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, 126 personnels supplémentaires pour la protection judiciaire de la jeunesse, dont 107 éducateurs. Ce plan de recrutement est au coeur de la justice de proximité que j'appelle de mes voeux, une justice proche, humaine, qui a le souci des plus faibles ; une justice qui garantit le respect du droit dans la vie quotidienne, car elle sera plus et de qualité ; une justice accessible pour tous les justiciables ; une justice de proximité non seulement pénale, mais également civile. sont les objectifs profonds de la justice de proximité. Pour la mettre en oeuvre, le projet de budget nous permet de disposer de moyens inédits, soit 200 millions d'euros, le fléchage de 1 100 emplois sur les 2 450 que je viens de vous présenter. Très concrètement, nous consacrerons 13 millions d'euros pour favoriser le recours à des magistrats honoraires et des magistrats à titre temporaire 28 millions d'euros pour la mobilisation accrue des délégués du procureur ; 20 millions d'euros pour la création de nouvelles unités médico-légales d'assistance de proximité aux victimes 79 millions d'euros d'augmentation des autres frais de justice pour renforcer les moyens d'investigation et donc l'efficacité de la justice. 20 millions d'euros au milieu associatif de la protection judiciaire de la jeunesse, pour renforcer la prise en charge rapide des délits du quotidien. Enfin, madame la sénatrice Boyer, nous prévoyons 10 millions d'euros pour le développement des bracelets électroniques et anti-rapprochement, le développement des travaux d'intérêt général et du travail non rémunéré, et pour le fonctionnement courant. Ces crédits et renforts supplémentaires sont particulièrement bienvenus dans le contexte actuel. Ce sont des moyens en plus pour le renseignement pénitentiaire, pour la réalisation de places dédiées aux détenus radicalisés, pour le recrutement et la formation d'agents spécialisés. Ce budget permet donc de répondre aux inquiétudes ou aux alertes exprimées par M. le rapporteur pour avis Marc, ou encore M. le sénateur Sueur.

495 places seront dédiées aux détenus radicalisés dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation, les quartiers de prise en charge de la radicalisation ou encore dans les quartiers d'isolement. une hausse des moyens de 10 %, seront consacrés à l'amélioration de la sécurité pénitentiaire pour accompagner le renforcement de la vidéosurveillance, lutter contre les drones malveillants ou encore déployer des systèmes de brouillage des communications. La surpopulation carcérale est une préoccupation majeure. Elle pose des défis en termes de dignité pour les détenus, de capacité à la réinsertion

Pour faire face à cette situation, mon action au sein du Gouvernement est double : développer les aménagements de peine les travaux d'intérêt général ou le développement de la surveillance électronique,

pour trouver le foncier nécessaire au lancement des 8 000 futures places d'ici la fin du quinquennat, mais, pour ce programme, j'ai besoin du soutien de tous les élus, et de vous particulièrement, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, pour convaincre les élus qui ont parfois quelques réticences à vouloir construire des établissements pénitentiaires sur leur territoire. Madame la rapporteure pour avis Vérien, monsieur le sénateur Bonnecarrère, vous avez appelé mon attention sur la rénovation numérique

en mode projet. Les services du ministère s'y emploient. À titre d'illustration, je peux vous citer trois grandes réalisations en 2021 le système d'information de l'aide juridictionnelle (SIAJ), le portail des agents et des détenus pour lequel une expérimentation est prévue à partir de mars 2021 en vue d'une généralisation dès la fin de l'année enfin, le portail des juridictions, qui remplacera progressivement les huit systèmes d'information du domaine civil utilisés dans les tribunaux judiciaires pour une procédure civile enfin dématérialisée.

Cet intérêt fait clairement écho à l'attente forte des justiciables, des avocats et de l'ensemble des métiers du droit en la matière. C'est la raison pour laquelle, le

c'est bien pour laisser du temps à la concertation en septembre et en octobre que nous avons été contraints d'introduire cette réforme par amendement au projet de loi de finances. Au total, ce sont donc 50 millions qui sont d'ores et déjà mis sur la table dès le 1janvier 2021 avec deux objectifs complémentaires : d'un côté, la hausse substantielle de la rémunération de l'heure travaillée par chaque avocat au titre de l'aide juridictionnelle et ce, je le redis, dès le 1janvier 2021, soit une hausse de 2 euros de l'unité de valeur une révision du barème, notamment pour mieux rémunérer les médiations ou l'assistance éducative. Il faut également pouvoir utiliser cet effort budgétaire comme moyen de levier pour développer les modes alternatifs de règlement des différends. d'une première marche de 50 millions d'euros. C'est un réel gage de crédibilité donné à la profession pour enclencher le nécessaire travail de fond sur l'avenir du métier d'avocat. Avec 50 millions d'euros supplémentaires, soit une augmentation de 7 % en crédits de paiement, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) n'est pas oubliée, notamment dans la perspective de l'entrée en vigueur le 31 mars prochain du code de justice pénale des mineurs, sur lequel l'Assemblée nationale a justement commencé à débattre ces jours derniers. Nous mettons les moyens pour permettre la mise en oeuvre de cette réforme : 72 magistrats, 100 greffiers spécialement dédiés sont mobilisés avec, en outre, la création de 252 emplois nouveaux à la protection judiciaire de la jeunesse entre 2018 et 2022. Plus globalement, les crédits supplémentaires alloués à la PJJ permettront de développer les alternatives aux poursuites dans le secteur associatif habilité et apporter une réponse plus rapide plus efficace à tous les actes de délinquance. Ils permettront également, madame la rapporteure pour avis Carrère, de poursuivre la politique de construction de vingt centres éducatifs fermés. Enfin, pour les personnels du ministère, j'ai décidé de mettre en oeuvre une politique de ressources humaines ambitieuse. Nous devons améliorer le fonctionnement de notre justice, en général. C'est le sens de ce projet de budget, qui s'en donne les moyens pour la première fois en plus d'un quart de siècle. Tous les maillons de la chaîne judiciaire seront renforcés avec le même objectif

Malheureusement, les crédits qui lui sont alloués souffrent d'un sous-financement chronique. Ce phénomène a d'ailleurs été dénoncé par le rapport Perben de 2020, qui a dévoilé que, en moyenne, le montant accordé à l'aide juridictionnelle est de en Europe lorsque nous n'investissons que 5,06 euros par habitant. Cette situation est inacceptable : la justice n'est pas un luxe et devrait être accessible à chacun de nos concitoyens, pas seulement à ceux qui ont les moyens de payer leurs frais judiciaires. Nous notons que le Gouvernement semble avoir compris la nécessité d'agir en la matière. En atteste l'augmentation de 49,7 millions d'euros dont a pu bénéficier l'aide juridictionnelle dans ce projet

qu'une rallonge de 53 millions d'euros est nécessaire, afin que la France puisse atteindre des standards similaires à ceux de ses partenaires européens.

Bien que le seuil de ressources pour en bénéficier soit extrêmement bas, nous le savons, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter sans que, dans le même temps, l'indemnisation des avocats ait été revalorisée.

Or, dans le contexte de crise sanitaire, sociale et économique que nous connaissons et d'une hausse très importante de la précarité, il est indispensable que chacun puisse avoir accès à la justice et défendre ses droits. Cet amendement vise donc également

mais, concernant les créations de postes, nous restons au-dessous du niveau nécessaire. Vous avez vous-même indiqué vouloir renforcer la justice de proximité mais, ce que vous n'avez pas précisé dans votre propos, c'est que vous parliez d'une justice pénale de proximité.

titulaires et, ainsi, d'améliorer la justice de proximité, notamment la justice civile de proximité.

et sociale d'une personne, et à informer le magistrat des mesures propres à favoriser ou à maintenir son insertion sociale. En raison de l'augmentation du nombre d'enquêtes qui, selon certaines estimations de la direction des affaires criminelles et des grâces, devrait passer de 80 000 en 2019 à 300 000 en 2021,

et jugement des affaires pénales, du programme 166, « Justice judiciaire ». Cette hausse serait compensée par une diminution des crédits de l'action n° 04, Gestion de l'administration centrale, du programme 310, « Conduite et pilotage de la politique de la justice », au regard des règles de dépôt des amendements en loi de finances.

également appelées enquêtes de personnalité présentencielles. Les ESR sont définies par le code de procédure pénale comme des investigations visant à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne et à informer le magistrat des mesures propres à favoriser ou à maintenir son insertion sociale.

à réévaluer la tarification des enquêtes sociales rapides, également appelées enquêtes de personnalité présentencielles. Les ESR sont définies par le code de procédure pénale comme des investigations visant à vérifier la situation matérielle,

Les associations ne le comprendraient pas, et ce d'autant plus, monsieur le ministre, que la direction des affaires criminelles et des grâces a estimé que le nombre d'enquêtes de ce type devrait passer de 80 000

la délégation aux droits des femmes du Sénat pointait les dysfonctionnements de la chaîne pénale. Parmi les solutions envisagées pour les pallier, les rapporteurs plaidaient pour la mise en place de permanences des juges aux affaires familiales le week-end, comme c'est le cas pour les procureurs, d'autant que la récente loi visant à agir contre les violences faites aux femmes prévoit désormais un délai maximum de six jours pour délivrer une ordonnance de protection.

sein de notre appareil judiciaire dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19. Les manques sont multiples : financier, matériel, en termes d'infrastructures et de personnels, etc. Cette situation dramatique entraîne non seulement une moindre capacité d'action de nos tribunaux judiciaires, mais surtout un service de qualité toujours déclinante, tant pour les usagers que pour les professionnels du droit. Alors que la grande majorité du contentieux civil a été mise à l'arrêt entre mars et juin, il est à craindre que l'engorgement massif des tribunaux ne soit de mise en en 2021, et ce d'autant plus qu'un ralentissement du traitement des affaires judiciaires se produira immanquablement à la suite de ce deuxième confinement.

que les 164 tribunaux judiciaires que compte le territoire national puissent bénéficier d'une dotation exceptionnelle de 100 000 euros.

prévu de créer que 40 nouveaux emplois pour l'encadrement et l'accompagnement des jeunes délinquants. Il va sans dire que cet effort est bien insuffisant dans la mesure où, dans le même temps, vous prévoyez l'ouverture de 105 nouveaux centres éducatifs fermés. Les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne sont, par principe, pas favorables à l'enfermement des mineurs délinquants, qui doivent être éduqués, réhabilités plutôt que punis et réprimés.

Ce bracelet constitue un outil de protection des victimes de violences conjugales, qui a fait ses preuves dans plusieurs pays européens. D'ailleurs, nous nous sommes calqués sur le dispositif espagnol, sachant que l'Espagne a consacré 6 millions d'euros par an à la mise en place de ce dispositif. Tout à l'heure, certains chiffres ont été annoncés. Je rappelle simplement que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, c'est-à-dire l'année dernière, le Gouvernement s'était engagé à ce que les crédits dédiés aux bracelets électroniques atteignent 5 millions d'euros dès leur déploiement en année pleine.

consacre 62,6 millions d'euros en autorisations d'engagement et 63,7 millions d'euros en crédits de paiement à la sécurisation des établissements pénitentiaires. Je rappelle que, en 2018, un rapport de la mission d'information relative au régime juridique des fouilles en détention a montré que la problématique des fouilles posait la question plus générale de la sécurité en détention et des moyens dont disposent les chefs d'établissement et les surveillants pour lutter contre l'entrée d'objets dangereux et illicites. La mission d'information proposait notamment de renforcer les moyens de contrôle des détenus en développant un contrôle renforcé l'aide d'unités cynotechniques.

pour 2021 prévoit déjà la création de 1 500 emplois, soit 240 emplois au-delà de ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice, dont 150 emplois pour renforcer l'équipe autour du magistrat. En outre, 50 postes de magistrats sont créés en 2021.

afin, notamment, de remédier à la carence en matériels. Les crédits de paiement du programme 166, « Justice judiciaire », s'élèvent à 3,7 milliards d'euros pour 2021, soit une augmentation de 208 millions d'euros par rapport à 2020. Les moyens de fonctionnement augmenteraient ainsi de 10 millions d'euros, afin d'adapter les modes d'organisation judiciaires aux enjeux numériques,

en lien avec les départements, contre une économie de 83 emplois liée à la restructuration des dispositifs de prise en charge. Ainsi, ce sont 84 emplois qui sont d'ores et déjà prévus au titre de la prise en charge éducative en milieu ouvert. Ce volontarisme affiché en termes de recrutement

Une projection de 1 000 BAR est prévue à l'issue de la première année de fonctionnement. La dotation prévue pour assurer le financement de la mesure s'élève à 4,7 millions d'euros en 2021. Elle sera complétée par une contribution du fonds pour la transformation de l'action publique à hauteur de 2,7 millions d'euros. L'augmentation des crédits

50 millions d'euros de plus qui lui sont consacrés. Cet effort permettra de financer les effets progressifs d'une nouvelle revalorisation des rétributions versées aux avocats, à hauteur de 50 millions d'euros par an en régime permanent. La moitié de cet effort est affectée à une revalorisation du montant de l'unité de valeur, qui passe de 32 à 34 euros, et l'autre moitié à une revalorisation ciblée du barème de rétribution, afin, notamment, de mieux indemniser le recours à la médiation.

L'amendement déposé par le Gouvernement pour revaloriser le montant de l'unité de valeur a en outre introduit une réforme de la commission d'office, afin de sécuriser la rétribution des avocats commis d'office lorsqu'ils interviennent en urgence, sans garantie de pouvoir être rétribués par le client. Il s'agit, j'y insiste, d'une première étape solide, tangible, crédible, qui doit permettre d'enclencher un processus essentiel

Les effectifs de magistrats et de fonctionnaires recrutés en 2021, ayant à suivre une scolarité de 31 mois pour les magistrats, de 18 mois pour les fonctionnaires de greffe, ne seront pas affectés en juridiction immédiatement. Ce que j'ai décidé, après m'être rendu en juridiction à la suite de ma nomination, c'est qu'il fallait au plus vite combler les vacances de postes parmi les agents de greffe. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la justice de proximité, j'ai proposé un recrutement exceptionnel de personnels contractuels qualifiés, très rapidement mobilisables,

Pour les services judiciaires, l'impact de la généralisation des ESR avoisine 1,55 million d'euros et pourrait être absorbé par l'augmentation significative des moyens alloués à l'action n° 02, Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales, du programme 166, « Justice judiciaire ». La mobilisation nécessairement accrue des associations qui mènent ces enquêtes sociales rapides m'a conduit

la justice de proximité, déclinée au civil et au pénal- et je n'oublie pas le civil -, est une priorité de mon ministère et des moyens massifs ont été obtenus. Je les rappelle : 914 emplois de contractuels, 13,1 millions d'euros pour favoriser le recours à des magistrats honoraires, à des magistrats à titre temporaire, et ainsi atteindre la limite maximale de 300 vacations 28 millions d'euros au titre de la mobilisation accrue des délégués du procureur, qui sont payés sur frais de justice ; 4 millions d'euros pour le fonctionnement courant correspondant aux créations d'emplois. Les moyens déployés pour renforcer la justice de proximité sont donc extrêmement importants et ambitieux.

dans les juridictions afin de rendre possible le travail à distance pour les activités prévues dans le plan de continuité d'activité, le fameux PCA. Depuis la reprise, 3 500 nouveaux postes ont été commandés ; leur distribution a commencé au mois d'octobre 2020.

C'est la fierté de la Chancellerie, et ma fierté, d'avoir demandé à la justice de poursuivre son oeuvre dans ces temps difficiles. Deux raisons à cela, madame la sénatrice

Le choix d'intégrer ce dispositif au sein de la plateforme technique de la surveillance électronique a permis à l'État de bénéficier d'une mutualisation des moyens et de sécuriser son calendrier prévisionnel de déploiement à la fin du mois de septembre 2020. À partir de 2021, la dépense récurrente devrait s'établir à 7,4 millions d'euros par an pour 1 000 mesures actives, en moyenne, sur l'année : 4,2 millions d'euros pour la téléassistance et la location des équipements et 3,2 millions d'euros pour le système d'information.

en quatre ans et de 9,6 % entre 2020 et 2021. Les crédits permettent de financer, notamment, la poursuite de la rénovation de la vidéosurveillance, avec la sécurisation périmétrique des établissements, lutte contre les drones malveillants ou encore le déploiement de systèmes de brouillage des communications illicites. Si l'on ajoute les crédits en faveur du renseignement pénitentiaire- 5,9 millions d'euros -, l'enveloppe globale atteint près de 70 millions S'agissant plus particulièrement du développement des unités cynotechniques, la première d'entre elles au sein de l'administration pénitentiaire a été créée en 2006 dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, permettant de disposer de moyens efficaces de recherche de produits stupéfiants, de monnaie fiduciaire, d'armes, de munitions ou de substances explosives. Deux nouvelles bases ont ensuite été mises en place : l'une à Toulouse en 2011 et l'autre à Lyon en 2015. Une quatrième base est en cours de création à Rennes. Le choix du terrain a été arrêté voilà quelques mois et les études de programmation sont en voie de finalisation, pour un lancement du concours

et qui annonçaient bien évidemment le déploiement en année pleine, n'ont pas été respectés. Pendant ce temps, des femmes meurent ! Exactement ! Il est donc important de voter ces crédits

dénoncent les violences qu'elles subissent, elles ont besoin d'être crues et prises au sérieux. Créer un cadre bienveillant et protecteur est indispensable pour permettre aux victimes de signaler les faits. Il s'agit de mettre fin à la culture du doute, qui prévaut souvent,

des victimes. Les unités médico-judiciaires, ou UMJ, assurent, sur demande de la justice, les examens médico-légaux des personnes majeures ou mineures victimes de violences. La finalité de l'examen est la rédaction d'un certificat médical descriptif des lésions physiques ou du retentissement psychologique, avec la détermination d'une incapacité totale de travail, ou ITT, au sens pénal. Pourtant le Grevio, le Groupe d'experts sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique,

tels que des infirmières spécialisées, par département et la conservation d'éléments de preuve, même si la victime ne souhaite pas porter plainte, en tout cas dans un premier temps. Quel

Et alors ? Il semble que le Premier ministre a dû vous rappeler qu'il ne fallait pas mélanger votre passé d'avocat et votre présent de ministre de la justice. Lors de ce procès,

qui aiment le pouvoir, il y a des femmes qui aiment le pouvoir : c'est comme ça. » Vous traitiez les parties civiles de « manipulatrices

! La société doit exercer un contrôle sur l'agresseur en recourant aux différents outils judiciaires de protection des femmes victimes de violences conjugales. Aucune violence révélée, et ce dès les premiers faits de violence, ne doit rester sans réponse pénale. Les outils judiciaires de protection existent, comme l'éviction du domicile du partenaire- ou

S'il se félicite des lois votées par le Parlement, il déplore le manque de moyens permettant de vérifier que ces nouvelles dispositions sont correctement appliquées. Il considère par exemple que « beaucoup de magistrats n'ont pas encore pris en compte l'importance de ce sujet, malgré les formations ». C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à attribuer davantage de moyens à la formation des magistrats, notamment pour créer des modules de formation continue relatifs aux violences conjugales. Dans le rapport qu'il a consacré à cette question, le HCEfh pointe la nécessité d'une telle formation.

Dans l'affaire Obiang- il s'agit du vice-président de la Guinée équatoriale -, le tribunal de Paris a conclu qu'« il serait moralement injustifié pour l'État,

qui sont, dans leur très grande majorité, éligibles à l'aide juridictionnelle (AJ). Toutefois, en raison de la nécessité d'un examen de cette éligibilité par les bureaux d'aide juridictionnelle (BAJ), les délais de rétribution des avocats souffrent d'un allongement considérable.

introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale pour certains contentieux à Paris est fort bienvenu : c'est pourquoi nous proposons de l'étendre aux procédures introduites devant le tribunal administratif, relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté, de liberté, sans préjudice du recouvrement par les bureaux d'aide juridictionnelle des sommes dont auraient bénéficié les personnes non éligibles. Cette mesure nous apparaît d'autant plus nécessaire qu'elle permettra, dans le même temps, un réel gain d'efficacité pour l'examen des demandes transmises aux BAJ dans le cadre d'autres contentieux. monsieur le rapporteur

Par ailleurs, cet amendement, en ce qu'il tend à prévoir des contrôles, ne remet pas en cause le principe posé par la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, qui reste inchangé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est conditionné au respect des conditions d'éligibilité, en particulier de celles qui concernent les ressources. Cette mesure vient donc utilement compléter le cadre posé par le Gouvernement. Les procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers, lorsqu'elles s'accompagnent d'une mesure restrictive de liberté, sont jugées en quatre-vingt-seize heures et ce sont les libertés des personnes concernées qui sont en jeu. Cet élargissement du dispositif dans un objectif de simplification administrative de bon aloi

Il dresse ainsi la liste des différentes procédures à l'occasion desquelles l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris dans l'hypothèse où la personne qu'il assiste ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'AJ. Si l'instauration d'une aide juridictionnelle garantie constitue une avancée dont nous nous réjouissons, la liste limitative proposée par le Gouvernement ne nous paraît pas suffisante. Cet amendement vise donc à y ajouter les désignations à l'audience et les désignations en urgence. L'amendement n°

? Ces amendements visent à ajouter à la liste l'assistance à la victime d'une infraction lors d'une audition par l'OPJ et la commission d'office d'un avocat par le bâtonnier ou par le président de l'audience de jugement, sauf pour les comparutions sur reconnaissance

À la différence du nouveau dispositif proposé par le Gouvernement, ceux-ci ne sont en effet pas compatibles avec le principe posé par la loi de 1991 selon lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle est conditionné au respect des conditions d'éligibilité.

Pour autant, plusieurs défis techniques sous-tendent ce dispositif, liés, notamment, à l'exigence de performances informatiques dont chacun ici saisit bien l'enjeu. C'est la raison pour laquelle notre assemblée avait adopté en juin dernier le report de huit mois de la mise en place de la Junip, la création doit donc intervenir au 1 septembre 2021. Comme le souligne le rapport de la rapporteure pour avis de l'Assemblée nationale consacrée à la transformation numérique de la justice, la Junip doit s'accompagner du développement d'un applicatif numérique natif,

devait initialement être créée au 1 janvier 2021. La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a repoussé cette date au 1 septembre 2021. Cet amendement vise désormais son report au 1 septembre 2022.

On ne peut maintenir une telle situation, qui créerait une dangereuse insécurité juridique, dans la mesure où les autres tribunaux judiciaires risqueraient de ne plus pouvoir ordonner des injonctions de payer, alors même que l'instance unique, la Junip, ne serait pas opérationnelle. Ce serait autant de contentieux de l'impayé qui retomberaient, sous forme de procédures contradictoires, dans le contentieux des tribunaux judiciaires, qui ont déjà beaucoup de travail- encore un doux euphémisme. Le traitement des contentieux de l'impayé selon la procédure contradictoire nécessiterait la mobilisation massive d'emplois supplémentaires, évaluée à

Il y a donc lieu de permettre une évaluation du dispositif envisagé, en concertation avec le Parlement, et de reporter la création de la Junip au 1 septembre 2022. Je me permets d'insister, de la façon la plus solennelle,

conduirait à un vide juridique qui causerait un grand tort à tous les secteurs de l'économie, notamment aux plus petites entreprises. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu'être éminemment favorable à cet amendement.

Merci